La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 19 avril 2018 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté.

Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je vous rappelle que l'auteur de la demande du débat disposera d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répondra pour une durée équivalente.

Dans un contexte international instable, nos concitoyens attendent de l'Union européenne qu'elle contribue à assurer leur protection effective.

Nous l'avons rappelé ici même, juste après les dramatiques attentats de janvier 2015. Nos propositions avaient été partagées par nos collègues de plusieurs États membres, également durement touchés par le terrorisme, lors d'une réunion interparlementaire tenue au Sénat sous la présidence de Gérard Larcher.

qui a permis de démanteler, le 26 avril dernier, des outils de propagande de Daech. EUROPOL s'investit aussi beaucoup dans les échanges d'informations, notamment grâce à son système SIENA,

Madame la ministre, peut-on escompter des progrès dans ce domaine ? Avez-vous des échanges avec vos homologues européens sur ce point précis ? Nous avons aussi besoin d'un parquet européen compétent pour lutter contre le terrorisme et la criminalité.

? La cybercriminalité représente une menace croissante. Les dommages ne sont pas seulement économiques, mais aussi politiques. EUROPOL s'est doté d'un centre de lutte contre la cybercriminalité. Il est souhaitable que chacun des États membres en fasse autant d'ici à 2019. La France dispose déjà d'une Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. L'Union européenne doit également contribuer davantage à la sécurité extérieure. En combattant les groupes terroristes au Sahel, nos soldats engagés dans l'opération Barkhane défendent l'ensemble de l'Europe. Le président Larcher leur a témoigné directement le soutien du Sénat lors de sa récente visite au Tchad et au Niger. Nous sommes en droit d'attendre un soutien plus important de nos partenaires européens. Nous devons progresser vers une Europe de la défense, complémentaire de l'OTAN. Nous devons aller vers une mutualisation des moyens, vers une interopérabilité, vers une action commune en matière de recherche et de développement et vers un rapprochement de nos industries de défense. C'est pourquoi nous appuyons le lancement d'une coopération structurée permanente entre vingt-cinq États membres, la mise en place d'un « fonds européen de défense » et celle d'un « Schengen militaire La Commission européenne propose aussi, pour la prochaine programmation budgétaire, un effort significatif avec un fonds de défense doté de 13 milliards d'euros afin de compléter les dépenses nationales en matière de recherche et de développement des capacités. Il nous semble nécessaire d'aller beaucoup plus loin sur le volet opérationnel. Les Européens doivent conduire ensemble des opérations militaires. À cet égard, madame la ministre, pouvez-vous nous donner des précisions sur le projet de force d'intervention européenne

est essentielle. Le défi migratoire est un autre sujet de préoccupation de nos concitoyens. Ils attendent des réponses de l'Union européenne. Il faut impérativement assurer la protection des frontières extérieures. Face à l'ampleur du défi, nous assistons enfin à une prise de conscience- certes tardive -de l'Union qui s'est traduite par le renforcement des moyens budgétaires et humains de l'agence FRONTEX.

conduit son action. Qu'en est-il de l'accès aux bases de données, instrument indispensable pour que cette action soit opérationnelle ? Qu'en est-il de la possibilité pour l'agence d'intervenir de façon quasi automatique dans un État qui serait défaillant pour assurer la protection effective de sa portion de frontière extérieure ? Qu'en est-il des procédures de retour groupé ? La refonte du système d'asile est un autre enjeu majeur. Les discussions se poursuivent au Conseil sur la réforme du règlement dit de Dublin qui précise les responsabilités des États membres dans le traitement des demandes d'asile. La question des relocalisations est particulièrement délicate. Elle a suscité de vives controverses entre États membres. C'est la solidarité européenne qui est en jeu. Un compromis est-il envisageable ? Nous souhaiterions connaître votre analyse sur ce point, Il faut aussi avancer dans la coopération avec les pays d'origine et de transit et avoir un plan ambitieux pour le développement de l'Afrique qui conditionne notre sécurité et la régulation des flux migratoires.

comme nous le souhaitions, un effort financier fortement accru sur les questions de sécurité, de migrations et de frontières.

et défend ». S'agissant de la sécurité, l'Union européenne reste très mobilisée face à la menace terroriste, comme le montrent les nombreux chantiers législatifs engagés pour mieux contrôler l'espace européen. L'urgence est donc maintenant de mettre pleinement en oeuvre l'ensemble des mesures prises et de les généraliser. Je pense d'abord à cette avancée majeure qu'est le PNR européen, qui doit être transposé dans tous les pays d'ici au 25 mai prochain.

Nous mettons également la pression sur la Commission et sur nos partenaires pour que le système d'entrées-sorties prévu pour les ressortissants des États tiers puisse être rapidement élargi aux ressortissants européens. Nous poursuivons la lutte contre le financement du terrorisme. Nous allons agir avec la Commission pour mieux contrôler les substances pouvant servir à confectionner des explosifs et mieux sécuriser les documents officiels. ailleurs, il est fondamental de mieux lutter contre la radicalisation sur internet. Nous encourageons la Commission à aller au-delà d'une approche centrée sur la contribution volontaire des acteurs du numérique à une autorégulation et à prévoir la mise en place de moyens contraignants pour améliorer la détection automatique et la suppression des contenus illégaux. S'agissant des outils européens dont nous disposons, vous avez évoqué la mise en place du parquet européen que nous avons soutenue depuis le début. Nous appuyons l'idée d'élargir sa compétence, au-delà des questions financières, à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontalière et au terrorisme. La Commission, je le crois, nous entend. Un mot enfin sur EUROPOL, qui joue un rôle irremplaçable pour le partage des informations. Ses compétences peuvent être utilisées de façon offensive, comme fin avril- vous l'avez rappelé, monsieur le président -contre les outils de propagande de Daech. Nous devons y avoir pleinement recours. Pour y jouer tout notre rôle, nous devons d'ailleurs veiller à y renforcer notre présence. J'ai eu de premiers échanges sur ces sujets avec la nouvelle directrice exécutive d'EUROPOL, Catherine de Bolle, avant même sa prise de fonctions. Enfin, je ne fais que le mentionner, mais peut-être y reviendrons-nous au cours du débat, gardons à l'esprit le développement de l'Europe de la défense, et en particulier le programme de développement de l'industrie de défense, précurseur du futur Fonds européen de défense en cours d'adoption et qui constitue une avancée majeure. Vous m'avez interrogée sur l'initiative européenne d'intervention. Ce projet que nous portons, et que le Président de la République avait annoncé dès le discours de la Sorbonne,

mieux programmer, mieux planifier, mieux partager nos évaluations sur la nature de la menace et sur la connaissance des théâtres autour des capacités françaises

J'en viens aux questions de migrations et de frontières. Le Gouvernement vous rejoint, monsieur le président, pour souligner toute l'importance du nouveau corps européen de gardes-frontières et gardes-côtes qui dispose de capacités nouvelles pour appuyer les États membres, qu'il s'agisse d'analyser les vulnérabilités des frontières externes, de participer à des reconduites à la frontière, ou d'agir en urgence, en cas de défaillance, à la demande du Conseil et avec l'accord de l'État membre concerné qui y a tout intérêt. La Commission propose, dans son projet de cadre financier pluriannuel, de porter le nombre de gardes-frontières et de gardes-côtes mobilisable au sein de la réserve d'intervention

Certains de nos partenaires paraissent relativement mal à l'aise avec cette partie précise de la proposition ambitieuse de la Commission et souhaiteraient plutôt un soutien accru aux gardes-côtes et aux gardes-frontières de chacun des États membres. Nous allons examiner cela en détail. Sur le plan interne- je pense à Schengen -, nous avons besoin de faciliter la possibilité de réintroduction des contrôles aux frontières internes lorsque le besoin s'en fait sentir, en particulier en raison de la menace terroriste. évidemment, une politique migratoire européenne ne peut réussir sans un partenariat renforcé avec les pays d'origine et de transit, en particulier en Afrique. La France a montré le chemin depuis le sommet restreint organisé à Versailles sur ce sujet en août 2017. Nous nous sommes dotés de moyens importants avec le Fonds fiduciaire d'urgence qu'il faut réabonder. Nous avons également mis en oeuvre un dialogue migratoire plus exigeant s'agissant des migrations économiques illégales et mis en place des dispositifs permettant de mieux protéger ceux qui peuvent prétendre au bénéfice de l'asile en veillant à éviter qu'ils ne risquent leur vie sur la route, en Libye comme en Méditerranée. Enfin, nous souhaitons que le Conseil européen de juin prochain permette de marquer des progrès sur la réforme du régime européen de l'asile. Les discussions restent très difficiles sur la révision du règlement de Dublin, en l'absence, qui plus est, d'un gouvernement italien de plein exercice. Nous soutenons les efforts de la présidence bulgare pour parvenir à la fois à un plus haut niveau de responsabilité des pays de première entrée, notamment dans le temps, et à un plus haut niveau de solidarité en encourageant des relocalisations volontaires en cas de crise et, si la situation est grave, en prévoyant un mécanisme automatique et contraignant de relocalisation. Nous y travaillons notamment avec nos partenaires allemands dans la perspective du Conseil européen de juin prochain. Je serai heureuse d'aborder ces points plus en détail, ainsi que les aspects que je n'ai pu évoquer, en répondant à vos questions. Mes chers collègues, chaque orateur dispose de deux minutes maximum pour présenter sa question avec une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente.

Ce nouvel article 42 fixe des objectifs en matière de connaissance des migrations climatiques et d'évolution de nos programmes d'aide publique au développement. Première occurrence des migrations climatiques dans le droit français, cette décision fera date. Si l'Europe a accueilli un million de migrants depuis 2015, elle n'a fait qu'effleurer la problématique à venir des migrations climatiques. Un récent rapport de la Banque mondiale, daté de mars 2018, indiquait ainsi que 143 millions de personnes seraient forcées de migrer sous l'effet du changement climatique d'ici à 2050. Le manque de nourriture, de ressources en eau, les canicules et les cyclones bouleverseront la géographie du monde tel que nous le connaissons. Des cadres internationaux existent déjà pour prévenir ces migrations. Le cadre de Sendai prévoit ainsi un effort collectif pour réduire les risques de catastrophes naturelles et prévenir les déplacements induits. Par ailleurs, les Nations unies ont mis en place un programme de réinstallation planifiée pour aider les migrants climatiques à s'installer et à rebâtir une nouvelle vie après leur exode forcé. Madame la ministre, selon la Banque mondiale, si des stratégies d'adaptation planifiées étaient rapidement mises en place sur la réduction des gaz à effet de serre ou sur l'anticipation des catastrophes naturelles,

alors que le solde migratoire est l'élément principal de la croissance démographique européenne à partir de 1990, nous pouvons affirmer que les conflits, les persécutions et les migrations sont devenus, depuis 2015, un défi pour l'Union. Sauver des vies, aider conjoncturellement les pays de transit importants à réduire les flux de migrants, l'enjeu est de taille et impose de faire preuve de pragmatisme : accord « un pour un », signé en mars 2016 avec la Turquie, permettant à 700 000 personnes de bénéficier

Je veux le dire avec solennité, sans verser dans l'angélisme, sans promettre ce que nous ne sommes pas en mesure d'assumer, nous avons un devoir d'humanité

Il est urgent de rappeler l'existence de nos frontières, non pas pour les transformer en barricades, en murs infranchissables, mais pour nous donner les moyens d'accueillir les migrants déracinés dans des conditions dignes. Personne ne peut accepter les conditions de vie des migrants, campant dans des parcs, devant des porches d'immeubles, sous des ponts du métro parisien, abandonnés et sans soutien. Nous devons être fermes avec les passeurs qui organisent sans vergogne le déplacement de femmes, d'enfants et d'hommes en mer Méditerranée, puis les laissent au hasard des chemins de montagne, sans le moindre respect. Nous devons être fermes avec ceux qui cherchent à se substituer à l'État, en organisant de façon empirique et médiatique un contrôle aux frontières. Madame la ministre, ma question est simple après le constat d'échec du règlement Dublin III, pouvez-vous nous assurer de la réalité d'une politique commune concernant la question migratoire, alliant fermeté et devoir d'humanité,

Nous devons aussi - et c'est ce que nous faisons - travailler avec les pays d'origine, pour mieux assurer le retour et la réadmission des migrants économiques illégaux. Nous le faisons avec des mesures incitatives, incitatives, notamment la mise en place de projets de développement, mais aussi dans la discrétion, bilatéralement, sans le porter sur la place publique, au cours de discussions avec chacun de ces pays, afin de nous assurer que les mesures de réadmission sont facilitées. Elles ont trop longtemps été rendues difficiles par des résistances et des obstacles. Nous le faisons entre pays membres de l'Union européenne et avec les pays d'immigration d'origine. Vous avez très justement cité, contre les passeurs et la nécessité d'augmenter encore notre coopération policière, au sein de l'Union européenne

Thani Mohamed Soilihi. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, selon un sondage d'Eurobaromètre réalisé auprès des citoyens européens en 2016, les deux problèmes les plus importants auxquels doit faire face l'Union européenne sont les migrations et la sécurité. Deux ans plus tard, ces thèmes sont toujours au coeur des préoccupations européennes. S'agissant des problèmes migratoires, l'Europe est confrontée depuis 2014 à une crise sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, conséquence directe de la multiplication des conflits armés, notamment en Syrie et en Libye. Le principal défi est de renforcer la solidarité européenne autour des thèmes des migrations et de la sécurité. Ces thèmes, Mayotte, région ultrapériphérique de l'Union européenne depuis 2014, les connaît bien, puisqu'ils ont constitué les principaux points de revendication de la vague de contestation qui a secoué l'île durant ces deux derniers mois. Ce département est soumis à une pression migratoire sans précédent et accuse une situation d'insécurité croissante. La pression migratoire exercée par les pays voisins sur le territoire mahorais, combinée à un taux de croissance démographique très élevé, pose des problèmes économiques et sociaux majeurs, comme l'ont montré les récentes tensions. Nous sommes face à une urgence, nécessitant une aide optimale de l'Union européenne dans la gestion durable des migrations, notamment par le biais de négociations devant aboutir à des accords internationaux et de partenariat avec les pays voisins. En effet, Mayotte connaît le taux de population en situation irrégulière le plus élevé de France, ce qui a pour conséquence directe la saturation de ses services publics, spécialement les écoles et les hôpitaux.

une dimension toute particulière, que le Gouvernement a pleinement à l'esprit. Je veux revenir sur les mesures inacceptables prises par les Comores le 21 mars dernier, pour interdire les reconduites de Comoriens entrés illégalement à Mayotte. Nous les avons publiquement Nous les avons publiquement condamnées, et nous sommes résolument engagés à les faire lever. Nous avons choisi de maintenir un canal de dialogue ferme et constructif avec les Comores, dans une logique d'engagement d'État à État, avec deux objectifs : lutter efficacement contre les filières d'immigration illégale et stabiliser à moyen terme la relation entre les Comores et Mayotte, ce qui doit passer par des actions ciblées sur les sources d'immigration irrégulière aux Comores, en particulier à Anjouan. Vous l'avez constaté, nous avons pris par ailleurs des mesures concernant les visas, qui concernent à la fois les passeports officiels comoriens et les demandes de visa sur passeport ordinaire. Il serait prématuré de dire que la situation a trouvé un règlement satisfaisant. Les ministres des affaires étrangères français et comoriens se sont entretenus le 19 avril dernier. Il n'y a pas encore d'accord concernant la réadmission, mais nous cherchons

Mayotte bénéficie en tant que région ultrapériphérique d'un soutien fort de l'Union européenne sur la période de budget actuel, 2014-2020. Ce sont ainsi 290 millions

Je souhaite mettre l'accent sur un programme de coopération transfrontalière entre Mayotte et les Comores, qui est financé à hauteur de 16 millions d'euros, pour développer les échanges commerciaux,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je suis intervenue récemment en faveur d'un jeune homme originaire du Darfour, au Soudan, pays qu'il avait fui à l'âge de douze ans

ce soit en Italie ou en France. Cette situation est loin d'être unique, vous le savez bien. Elle vient toutefois illustrer sans ambiguïté la nécessité, si l'on veut que le droit d'asile ait encore un sens, de revenir sur le règlement de Dublin. L'Union européenne ne s'y est pas trompée, et la Commission européenne s'est attelée à la refonte de ce règlement qui détermine l'État membre responsable de l'instruction d'une demande d'asile. En France, le Parlement examine en ce moment le projet de loi Asile et immigration, sans aucune considération pour les négociations et travaux en cours au niveau européen. Si ! Ma question est simple : de quelle manière le Gouvernement compte-t-il peser ? Quelles positions a-t-il l'intention de défendre au niveau européen,

Le règlement de Dublin a été adopté avant la vague migratoire de 2015. À l'évidence,

n'ont pas souhaité demander l'asile dans le pays dans lequel ils sont entrés. Madame, vous levez les yeux au ciel, mais lorsqu'on arrive du Soudan du Sud, on peut décider de faire du shopping de l'asile, et trouver qu'on est mieux en Suède qu'en Italie ! Comment osez-vous utiliser Italie ? Je suis allée au Soudan du Sud, et je vous invite à faire la différence entre ces pays et les pays européens.

européenne. Aujourd'hui, il faut renforcer la responsabilité des pays par lesquels les demandeurs d'asile entrent dans l'espace européen et la solidarité de l'ensemble de l'espace européen. De ce point de vue, la présidence bulgare du Conseil de l'Union européenne a fait une proposition que nous soutenons : il s'agit de traiter la situation, soit lorsqu'elle est normale, soit lorsqu'une crise migratoire commence, soit lorsque cette crise s'aggrave, avec des obligations de

ou obligatoire lorsque la crise s'aggrave. Aujourd'hui, l'Italie n'a pas un gouvernement en mesure de défendre une position. Nous attendons avec impatience la formation d'un nouveau gouvernement italien, pour essayer d'avancer sur une rénovation du règlement de Dublin.

Ce n'est pas un hasard si ce même point est mis en avant par l'ensemble de mes collègues. Vous avez d'ailleurs, par anticipation, répondu aux questions en évoquant votre souhait d'un plus haut niveau de responsabilité des pays de première entrée et d'un plus haut niveau de solidarité des pays dits « de deuxième ligne ». Vous avez dessiné des perspectives pour le mois de juin prochain. J'attends de votre part quelques précisions, pour que nous soyons certains de la volonté d'impulsion de notre gouvernement.

Toutefois, on l'a vu, les décisions de relocalisation n'ont pas été respectées par certains États membres. Aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de négocier une nouvelle révision du règlement de Dublin, les divisions au sein de l'Union européenne sont fortes.

des procédures, des délais et des critères utilisés dans l'Union européenne. De ce point de vue, le projet de loi Asile et immigration qui sera bientôt présenté à la Haute Assemblée va dans le sens de cette harmonisation.

Dans cette logique, les collectivités accueillant un nombre important de migrants devront être éligibles au fonds de cohésion. Ce serait un soutien

solidarité. Il est louable de proposer que les demandeurs d'asile puissent aller dans tous les pays de l'Union européenne. Mais quelles garanties avons-nous que les procédures seront les mêmes dans chaque pays ? Tel n'est pas le cas aujourd'hui ! Et les directives Procédure et Accueil ne suffisent pas, les procédures nationales étant aujourd'hui complètement divergentes. Comment faire pour arriver à une surveillance

notre pays a rempli ses obligations à la fois en matière de réinstallation depuis les pays extérieurs à l'Union européenne et de relocalisation, qu'il s'agisse de la Grèce,

de nouveaux engagements et mis en place, au Niger et au Tchad, une nouvelle procédure de réinstallation. Nous incitons nos partenaires européens à nous accompagner

au sein de la communauté européenne, les élus ne puissent pas se prononcer sur des plafonds et le choix des personnes à accueillir, en fonction de nos besoins et de notre

tant qu'il y aura autant d'inégalités entre les pays et aussi peu de perspectives d'éducation, de formation et d'emploi dans un certain nombre de pays du Sud, l'immigration illégale se poursuivra. La parole est

Comment aborder cette situation avec autant d'humanité que de réalisme ? Les solutions extrêmes, fermeture des frontières ou accueil de tous, ne sont pas réalistes.

certains pays ont apporté des restrictions à leur droit du sol. Êtes-vous ouverte à une évolution de notre droit en la matière, afin de refuser l'acquisition de la nationalité française à des enfants nés de parents en situation irrégulière ? La parole

plusieurs autres années au Maghreb. Depuis que je suis ministre chargée des affaires européennes, je me suis rendue à plusieurs reprises dans des camps de réfugiés et des foyers de mineurs isolés. Je crois donc que je sais de quoi je parle, parce que j'y suis allée voir de près, sans rester à l'abri de mes fonctions parisiennes. Monsieur le sénateur, vous parlez de chiffres français éloquents en matière d'arrivées de migrants et de demandeurs d'asile. Que devraient dire nos partenaires allemands, qui ont accueilli en 2015 plus d'un million Je voudrais le rappeler, puisque vous mettez en avant l'échelle européenne sur un sujet qui- vous le savez et, je crois, vous vous en réjouissez -est un sujet de compétence nationale propre, celui de l'acquisition de la nationalité. Il n'y a pas encore- et personne ne le souhaite -de politique communautaire en matière d'acquisition de la nationalité dans les États membres ; je ne vois donc pas très bien ce que l'Union européenne a à voir avec tout cela. J'ai le sentiment qu'on mélange beaucoup de choses à parler à la fois de demandeurs d'asile et d'acquisition de nationalité.

une connaissance suffisante de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, ainsi que l'adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République française. Ce n'est pas vrai ! Ce

Par conséquent, je m'étonne que le ministre des affaires européennes n'ait pas une vision globale de ce que peut être la politique de la France pour défendre ses intérêts au niveau au niveau européen. Votre réponse confirme celle que vous venez de faire à M. Pemezec. Décidément, nous sommes gouvernés par des technocrates ! Monsieur le président, madame la ministre, ce débat sur l'Union européenne face aux défis de la sécurité, des migrations et des frontières est attendu non seulement par nos compatriotes, mais aussi, en ce 9 mai, par tous les citoyens européens. Pourquoi ? ? Parce que nous avons face à nous une véritable bombe démographique. Selon les projections démographiques des Nations unies, la seule population de l'Afrique subsaharienne pourrait passer de 960 millions à 2 milliards d'habitants d'ici d'ici vingt-cinq ans. C'est naturellement considérable. Que l'on analyse la question à l'horizon de quelques semaines, de plusieurs années ou des prochaines décennies, le même constat s'impose plus que jamais, l'Europe va devoir apprendre à aborder cette question de l'immigration avec responsabilité, sous peine de voir nos démocraties submergées par le populisme. J'en viens à ma question, qui comporte plusieurs volets. Face à cette réalité démographique, peut-on réellement tenir le cap de la différenciation stricte- je sais que ce sujet est tabou -entre droit d'asile politique et immigration irrégulière, car économique ? En réalité, cela revient à accepter ceux qui meurent de peur et à repousser ceux qui meurent de faim. Cela revient surtout à nier que les véritables ressorts de l'immigration sont la misère, l'instabilité politique et l'absence de projet collectif. alors que la gravité de la question exigerait une politique européenne intégrée ambitieuse, comment articuler cette politique avec des politiques nationales qui, en la matière, restent extrêmement diverses ? Comment, aussi, articuler cette politique européenne de l'immigration avec celles des pays situés entre le Sahara et la Méditerranée- je veux parler des pays du Maghreb ? La parole

à l'occasion d'un conflit ou en raison de leur race, de leur religion, de leurs croyances politiques, de leurs orientations sexuelles, donc tous ceux qui relèvent de la convention de Genève,

par l'exil. Ce défi relève évidemment d'abord de la responsabilité des autorités de ces pays. Mais c'est aussi notre responsabilité de pays partenaire que de travailler, comme je le disais tout à l'heure,

quelle alternative avons-nous ? Si l'Afrique se développe, nous aurons un partenaire de croissance sur lequel nous pourrons nous appuyer. Si le destin de jeunes Sahéliens, en particulier, consiste nécessairement à aller chercher ailleurs qu'en Afrique, ici, en Europe, où nous ne pouvons pas tous les accueillir, on aura, en Afrique, de moins en moins de personnes qualifiées, de plus en plus de tensions, et donc de plus en plus de crises à gérer, car elles auront des conséquences sur notre sol.

l'Union pour la Méditerranée reste une bonne idée. Elle n'a d'ailleurs pas échoué sur ses objectifs, mais du fait des révolutions arabes et de la crise financière de 2008. Nous pensons donc qu'il est temps de réexplorer cette idée et de travailler à sa mise en oeuvre. La parole

Nous, sénateurs français, avions eu l'occasion d'analyser cet accord grâce aux travaux d'une mission d'information ayant pour objectif d'évaluer le bien-fondé et les conséquences de cette réponse, qui nous est apparue comme fragile, ambiguë et partielle face aux enjeux migratoires auxquels l'Europe a été et est confrontée. À l'aune des mutations politiques dangereuses que connaît la Turquie ces derniers mois, en particulier la reprise du conflit armé entre l'État et le parti du peuple kurde, le bien-fondé de cet accord sombre peu à peu. Pourtant, le 14 mars dernier, la Commission européenne dégageait une enveloppe supplémentaire de trois milliards d'euros destinée à aider la Turquie à accueillir les réfugiés syriens sur son sol. Cette seconde tranche d'aide montre qu'en dépit des tensions avec Ankara et des défauts de cet accord, ce dernier est encore mis en oeuvre. Bon nombre d'ONG et de personnalités politiques européennes ont appelé à une évaluation juridique de ce pacte. Cet accord serait en effet illégal parce qu'il reposerait sur le postulat erroné selon lequel la Turquie est un « pays tiers sûr ». Une clarification de la nature de la protection offerte dans un « pays tiers sûr » s'impose. Si nous nous résignons à accepter de sous-traiter le droit d'asile à des pays tiers, ceci doit être au minimum garanti par le caractère effectif de la protection, qui doit être identique à celle qui est accordée dans l'Union européenne- notamment à l'application du principe de non-refoulement. La Turquie présente-t-elle vraiment un haut niveau de garanties et de protection pour les demandeurs d'asile ? Le 25 avril dernier, les eurodéputés ont décidé de retirer la Turquie de la liste commune des pays d'origine sûrs. Mais, selon la Commission européenne, ce vote ne concerne pas l'accord bilatéral UE-Turquie, mais seulement les cas de nationaux turcs. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Peut-on penser que le retrait

est à Mme la ministre. Madame la sénatrice Gisèle Jourda, je voudrais rappeler que la déclaration Union européenne-Turquie de mars 2016 a permis que le nombre d'arrivées dans les îles grecques baisse de 97 et que le nombre de décès de migrants en mer Égée soit divisé par 10. Ce dispositif a permis de lutter efficacement contre les filières de passeurs ; nous sommes donc attachés à sa poursuite et à sa reconduction. Je rappelle aussi ce que je disais tout à l'heure : la Turquie est le pays au monde qui accueille le plus grand nombre de réfugiés. C'est un effort colossal,

indiquer que nous travaillons à la poursuite de notre coopération avec la Turquie en matière d'aide aux réfugiés. Ce que vous avez mentionné à propos du Parlement européen est une discussion : ce n'est en rien une décision. Je voudrais en outre préciser que que l'aide européenne versée au profit des réfugiés en Turquie l'est très majoritairement, presque exclusivement, à des acteurs non étatiques- collectivités locales, associations -qui viennent en aide à ces réfugiés et font un travail qui mérite d'être salué.

la présence dans notre tribune d'honneur de Mme Christine Defraigne, présidente du Sénat belge. Au nom du Sénat tout entier, je lui souhaite une cordiale bienvenue en cette journée de l'Europe. C'est aussi l'occasion pour moi de souligner l'excellence des relations d'amitié et de travail entre nos deux institutions. À l'issue de notre séance, Mme Defraigne aura un entretien avec le président Jean Bizet et le bureau de la commission des affaires européennes sur les grands sujets de l'actualité de l'Union européenne. Nous reprenons le

comme si l'on souhaitait traiter la question des frontières européennes et de l'immigration en catimini. Le 9 mai, c'est le 9 mai ! Une mésaventure qui m'est arrivée récemment renforce ma crainte en ce domaine. Rapporteur spécial de la mission budgétaire « Immigration, asile et intégration », j'avais souhaité me procurer un document signalé par la commission des affaires européennes « arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés lors de l'évaluation de 2016 de l'application, par la France, de l'acquis de Schengen dans dans le domaine de la gestion des frontières extérieures ». Ce document- vous aurez remarqué le magnifique jargon technocratique qui le caractérise -émane de l'Europe. Mon collaborateur s'étant vu refuser la consultation de ce document, je me suis moi-même rendu à la commission des affaires européennes, où l'on m'a signifié que j'avais le droit de le lire, mais non de le copier ou d'en emporter un exemplaire, comme s'il était normal de cacher aux parlementaires des recommandations de l'Union européenne à la France sur un sujet parfaitement régalien. Ma première question, madame la ministre, est donc la suivante : si l'on souhaite réconcilier les Français avec la politique et la construction européennes, ne pensez-vous pas qu'il serait légitime d'associer le peuple français et ses représentants aux débats fondamentaux portant sur notre sécurité, sur nos frontières et sur l'immigration ? Ma deuxième question a trait à ce que votre ministère a fait en réponse à la recommandation du Conseil européen dont je parlais à l'instant. Cette recommandation m'a en effet fait froid dans le dos. On y lit que, dans le port de Calais, les informations ne circulent pas bien d'une équipe à l'autre ; qu'à Roissy, les effectifs sont insuffisants pour assurer les vérifications aux frontières, et qu'il y manque du matériel adéquat ; qu'à Orly, les contrôles des membres d'équipage laissent à désirer. Il s'agit de la France Pourriez-vous nous dire, madame la ministre, si ces graves défauts relevés par le Conseil européen existaient réellement, ou s'ils n'étaient qu'imagination de technocrates bruxellois ? Et si ces défauts existaient bel et bien, qu'avez-vous mis en place pour remédier à cette situation préoccupante pour la sécurité des Français et pour l'identité de la France ? La

de notre pays. Je suis surprise que vous mettiez en avant le fait que la représentation nationale n'y soit pas associée ; c'est tout le contraire qui est vrai. S'agissant du document que vous mentionnez, à ma

Je m'engage devant vous à revenir sur cette question et à vous répondre lorsque la Commission européenne nous aura adressé son évaluation définitive.

à la crise migratoire. Il faut regarder ce qu'ont fait, en la matière, le Liban, la Turquie ou la Jordanie. La crise humanitaire n'est pas terminée en Syrie : d'autres vagues peuvent arriver. Or l'absence de résilience conduit l'ensemble des pays européens à envisager leurs relations avec leurs voisins, en particulier leurs voisins du Sud, d'abord

n'ira qu'en s'aggravant tant que nous ne changerons pas de paradigme, tant que nous considérerons que des régimes autoritaires à nos portes sont une garantie de surveillance des frontières de l'Union européenne. Madame la ministre, j'ai deux questions. D'une part,

La Jordanie a fait plus, la Turquie a fait plus, certes. Je vous rappelle quand même, madame la sénatrice Benbassa, que beaucoup de demandeurs d'asile ne souhaitaient pas venir en France à cause du niveau de chômage qui y prévalait, et préféraient partir en Allemagne ou en Suède. Je voudrais aussi indiquer que lorsqu'il s'agit d'un conflit comme le conflit syrien, il est assez habituel que les personnes fuyant une zone de guerre cherchent à rester à proximité, parce qu'elles ont l'espoir- et nous partageons cet espoir avec elles

Nous souhaitons clairement une amélioration de la délivrance des laissez-passer consulaires par les pays dont sont originaires des migrants économiques illégaux que nous voulons raccompagner. Nous menons ce dialogue avec l'ensemble de ces pays, comme le font aussi, bilatéralement, nos partenaires européens. Et la question de la délivrance de visas, en particulier de visas officiels,

de l'aide au développement européenne. Mais le Parlement européen contrôle l'aide au développement versée par l'Union européenne. Si vous avez, monsieur le sénateur, une question particulière et un souhait particulier s'agissant de ces questions de contrôle, je vous invite à me les communiquer et je vous répondrai par écrit. La

sur les problèmes d'immigration, on se demande si on est sur la même planète ! Dans la pratique, soit il s'agit de débats très techniques, et de modifications à la marge,

l'explosion démographique en Afrique, où voulez-vous qu'aillent les Africains, sinon par définition vers l'Europe ? Or je constate que le Parlement européen et la Commission européenne n'avancent pas d'un iota sur ce sujet.

l'effet du 9 mai, une fois par an ! Mais je vous promets que je ne le répéterai pas. Je voudrais tout de même vous rassurer : l'Union européenne est le premier donateur d'aide à l'Afrique. à l'Afrique. Pays membres et Union européenne confondus, ce sont 19 milliards d'euros d'aide au développement qui viennent d'Europe vers l'Afrique chaque année. S'agissant de l'aide plus spécifiquement destinée à lutter contre les migrations, le Fonds fiduciaire d'urgence atteint 3 milliards d'euros, et nous allons chercher à l'abonder de nouveau, tant avec des crédits

en direction des pays qui en ont le plus besoin, qui se trouvent au Sahel. Je n'ai parlé que d'aide au développement ; je n'ai pas parlé de notre action militaire, qui sert aussi à la stabilisation de cette partie de l'Afrique et à la lutte contre le djihadisme,

! La parole est à M. Cyril Pellevat. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dans le respect des accords de Schengen, plusieurs pays ont rétabli les contrôles à leurs frontières nationales : l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Suède, la Norvège, l'Italie, la République tchèque, la Slovaquie, la Belgique, la Pologne, Malte et la France. l'ont fait en raison de la crise migratoire ; nous l'avons fait pour contrer la menace terroriste à la suite des attentats du 13 novembre 2015. Mais la crise migratoire nous touche tout autant que les autres. L'Union européenne fait face à une crise sévère, qui nourrit d'ailleurs des mouvements populistes dans nombre de ses États membres. En 2017, les États membres de l'Union européenne ont accordé un statut protecteur à 538 000 demandeurs d'asile venant principalement de Syrie, d'Afghanistan et d'Irak. Les principaux pays ayant accordé un statut sont l'Allemagne, pour 60 % du total, la France, l'Italie, l'Autriche, la Suède, la Grèce, la Belgique et le Royaume-Uni. Face à la crise migratoire qui a commencé en 2015, l'Union européenne n'a pas toujours vu juste. Le système des a par exemple échoué. Il s'agissait de centres d'enregistrement des migrants destinés à répartir les nouveaux arrivants. L'Union européenne a été mise face à la faiblesse de sa politique d'immigration et d'asile. Selon vous, madame la ministre, quels sont les principaux impacts de cette crise migratoire ? crise migratoire ? Elle a connu son apogée en 2016, mais elle perdure. Rappelons que l'Union européenne, ce sont 500 millions d'habitants, dont 35 millions sont nés à l'extérieur des frontières, 20 millions sont étrangers et 1 million sans papiers. Les conflits, notamment en Syrie, perdurent. Les migrants venant d'Afrique sont très nombreux également. Les migrants économiques se mêlent aux réfugiés de guerre. Hormis le renforcement des contrôles aux frontières, l'une des solutions semble résider dans une meilleure coopération de l'Europe avec les pays tiers. Madame la ministre, pouvez-vous nous dire comment l'Union européenne entend renforcer la lutte contre l'immigration irrégulière ? La parole

ce nombre décroissait, il augmentait encore dans notre pays. Mais je voudrais apporter une indication qui me paraît aussi importante pour éclairer l'ensemble de notre débat : la première nationalité de demandeur d'asile, en France, en 2017, est la

contre les trafics d'êtres humains, sans lesquels ces personnes ne pourraient pas venir et rester sur notre territoire. Je voulais faire cette réponse, car je constate, à la lumière de l'ensemble des échanges que nous avons eus,

pour des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Nous savons aussi qu'un certain nombre de pays sont candidats à l'adhésion à l'Union européenne. Nous ne voyons jamais notre attractivité ; nous ne voyons que nos faiblesses. Nous avons regretté le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire signé avec l'Iran. Et, dans le concert des nations, peu nombreux sont ceux qui applaudissent. Ceux qui, comme nous, considèrent que l'accord reste valable

seule voix -de convaincre les uns et les autres de revenir à la table et de faire en sorte que l'accord nucléaire iranien, qui était un immense progrès dans la lutte contre la prolifération, puisse trouver un nouveau développement. Il serait tout de même paradoxal que l'Iran soit puni d'avoir respecté cet accord au moment où la Corée du Nord, qui, elle, est allée jusqu'au développement d'armes nucléaires, serait récompensée de n'avoir respecté aucun traité international. Vous avez évoqué la nécessité de bâtir une Europe de la défense. C'est précisément ce que nous faisons. On en a parlé pendant soixante ans sans rien faire ; depuis six mois, on en parle moins, mais on agit beaucoup plus. Je pense à la coopération structurée, à l'ébauche d'un fonds européen de défense et au projet français d'initiative européenne d'intervention, qui permettra demain

choqué. Étant un gaulliste frénétique, je considère que la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. Or j'ai entendu un certain nombre de ministres indiquer que le retrait de M. Trump créait un problème pour les entreprises françaises installées en Iran, celles-ci ayant triplé leur chiffre d'affaires depuis trois ans. Je le dis- avec tout le soutien que j'apporte aux entreprises françaises - : la France, ce ne sont pas les entreprises qui s'installent en Iran ; la France, c'est la paix, les droits de l'homme et la liberté

concitoyens. En matière de lutte contre le terrorisme, la création d'une Union de la sécurité et l'amélioration de l'alimentation, de l'utilisation et de l'interopérabilité des bases de données européennes sont essentielles.

national. La défense doit reposer sur une vision stratégique partagée, fondée sur une revue stratégique de la défense européenne. Le couple franco-allemand est essentiel.

pas d'entrer dans le jeu d'une politique de retour ne devrait plus être bénéficiaire d'une aide au développement. L'Europe est un grand pays, solidaire et généreux. Mais la générosité a des règles. Nous savons très bien qu'un certain nombre d'États, notamment africains, n'accordent des retours et des réintégrations que sur les doigts d'une seule main.

Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je vous rappelle que l'auteur de la demande du débat disposera d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répondra pour une durée équivalente.

Mais il doit d'abord être un atout pour les producteurs européens. Certes- et heureusement ! -, l'Europe n'a pas fait le choix du repli, dont les conséquences économiques seraient néfastes. Elle s'est ouverte sur le monde. Mais, en acceptant l'ouverture, elle doit aussi veiller à préserver ses intérêts économiques. Nous souhaitons en particulier que l'Union soit ferme et unie face aux initiatives américaines concernant l'aluminium et l'acier. Où en est-on des discussions avec les autorités américaines ?

d'une véritable stratégie industrielle européenne qui permettrait à notre continent de reconquérir le terrain perdu dans ce domaine. L'Europe doit rattraper son retard en matière d'investissement. Nous avons soutenu l'augmentation de la capacité et de la durée du Fonds européen pour les investissements stratégiques. La Commission européenne propose désormais de créer un d'investissement qui permettrait, par le jeu de garanties, de mobiliser 650 milliards d'euros d'investissements. Il faut parallèlement lever les obstacles réglementaires L'énergie doit être une priorité. L'Europe ne sera pas compétitive sans une énergie sécurisée, accessible et bon marché. Nous appuyons le projet d'une Union de l'énergie, tout en veillant à une bonne articulation entre les compétences de l'Union et celles des États membres. Pouvez-vous nous éclairer sur l'état des discussions en cours sur le paquet de textes présentés par la Commission européenne ?

L'innovation doit constituer une autre priorité. L'Europe peut apporter une réelle plus-value dans ce domaine. La Commission européenne propose un nouveau programme, intitulé, doté de 97,6 milliards d'euros, soit 53 % d'augmentation par rapport au cadre actuel. Elle souhaite afficher clairement la priorité accordée à l'innovation, avec un Conseil européen de l'innovation, qui constituerait un guichet unique en matière d'innovation de rupture. Quelle est l'appréciation du Gouvernement sur ces initiatives ? Personnellement, j'attire depuis quelque temps du Gouvernement sur deux points bien particuliers. D'une part, l'Europe n'est pas dotée de supercalculateurs de nouvelle génération alors que nos voisins d'outre-Atlantique et le bloc asiatique le sont.

pour la compétitivité européenne, l'Union économique et monétaire doit occuper une place centrale. C'est pourquoi son approfondissement doit demeurer une priorité. Dans le cadre du groupe de suivi sur la refondation, le Sénat avait formulé des propositions. Pour le prochain cadre financier, la Commission européenne prévoit un programme de soutien aux réformes, à hauteur de 25 milliards d'euros, et une fonction de stabilisation de l'investissement, avec une capacité de prêts de 30 milliards d'euros. Une feuille de route franco-allemande a été annoncée. Mais, à ce stade, on constate plutôt des divergences. Cela nous désole. Pouvez-vous nous rassurer sur une position commune de la France et de l'Allemagne d'ici au prochain sommet de la zone euro et au Conseil européen de fin juin ? L'Europe a pris conscience de son retard dans l'innovation et la régulation, mais également de sa faiblesse vis-à-vis des grands acteurs privés de l'internet. Face à des comportements contestables, comme l'optimisation fiscale ou l'abus de position dominante, les pouvoirs publics paraissent plus enclins à la fermeté. La Commission européenne a proposé une stratégie globale et ambitieuse. L'entrée en vigueur du règlement sur la protection des données personnelles doit être saluée. Et si l'Europe a eu un retard technologique important, elle a, je le crois, aujourd'hui ouvert une nouvelle porte, celle de l'éthique.

Le Sénat préconise de simplifier le déclenchement des mesures conservatoires, afin d'éviter que ne persistent des entorses aux règles de concurrence pendant la durée souvent très longue des procédures déclenchées par la Commission européenne.

les plateformes numériques structurantes pour l'économie, en leur appliquant notamment le principe de loyauté. Que peut-on attendre des propositions de la Commission européenne dans ce domaine ? Nous devons aussi parvenir à une taxation effective des revenus créés par l'activité numérique, en matière de fiscalité directe comme indirecte, avec une assiette rattachée au territoire de l'activité effectivement réalisée, que l'on appellerait « présence digitale significative ». Pouvez-vous éclairer

Mais le dispositif aurait au moins le mérite d'être enclenché dès maintenant. À l'ère numérique, le droit d'auteur et les droits voisins doivent être pérennisés par une assise

et la politique industrielle. Il faut soutenir la croissance des start-up européennes en Europe, en mobilisant les outils de financement et en levant les barrières à leur développement européen. L'Union européenne doit aussi défendre son ambition numérique dans les négociations commerciales

C'est la souveraineté proprement dite des États qui peut être mise à mal, de même que le développement d'une économie numérique, lequel ne peut que reposer sur la confiance de ses acteurs. La parole

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires européennes, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie tout d'abord de votre invitation. Nous le savons tous : le cadre européen est

Nous vivons une époque où les innovations structurantes, les évolutions techniques, les approches nouvelles en termes de production, de collaboration, de services ou de consommation s'accélèrent fortement et bouleversent non seulement les chaînes de valeur, mais aussi nos modes de vie. Ce qui est frappant également, c'est que l'origine de ces innovations se diversifie. Elles ne sont plus l'apanage des grandes puissances occidentales ni de grands groupes industriels historiquement établis. Il faut de plus en plus raisonner en dynamique, et anticiper plutôt que s'adapter. La compétitivité de l'Europe dans la durée repose largement sur sa capacité à intégrer les nouvelles technologies dans les produits de ses entreprises, dans les processus de production, dans leurs relations avec les clients et les partenaires. Dans la concurrence Dans la concurrence mondiale, notre continent a des atouts majeurs à faire valoir : une recherche de qualité, un tissu d'entreprises dynamiques, des têtes de filières qui créent de l'activité au sein de l'Union européenne, des compétences et des valeurs. Mais il faut aller plus loin si nous voulons que l'Union européenne joue pleinement son rôle de grande puissance économique mondiale au profit des citoyens européens. Nous devons définir et défendre une stratégie industrielle vraiment européenne, notamment sur l'innovation de rupture ; ce sera le premier thème de mon intervention. Nous devons aussi défendre nos valeurs, que ce soit en menant une politique commerciale ferme et sans naïveté ou en répondant aux défis posés par le développement des acteurs numériques ; ce sera le second thème de mon propos. La période est décisive, car nous devons prouver notre capacité à relever ces défis, en particulier avec le lancement des discussions sur le prochain budget européen, qui doit être à la hauteur des enjeux. nous devons bâtir une Europe de l'industrie, à la pointe de l'innovation de rupture. Face à la Chine ou aux États-Unis, une stratégie industrielle purement nationale n'a plus grand sens. Le Gouvernement entend bien pousser auprès de la Commission et de nos partenaires européens des initiatives ambitieuses et concrètes en matière de politique industrielle européenne. C'est à l'échelle européenne que nous pouvons créer des écosystèmes industriels de pointe et des « champions » capables de peser sur la scène mondiale. C'est aussi par l'Europe que pourra s'établir notre autonomie stratégique dans des technologies-clés : la cybersécurité, le véhicule autonome et connecté, l'aéronautique et l'espace, l'intelligence artificielle. L'Europe nous donne la force de frappe nécessaire pour mener de grands projets industriels intégrés, du laboratoire à l'usage : dans les supercalculateurs, par exemple, ou les nanotechnologies. En matière de R&D, l'Union européenne s'est dotée de bons instruments, mais ils concernent surtout l'innovation incrémentale. Les sujets complexes d'innovation radicale méritent une approche spécifique et un cadre fortement mutualisé en Europe. Notre puissance de feu en matière d'innovation de rupture est déterminante pour notre compétitivité. Elle repose sur des projets qu'on appelle « », c'est-à-dire très intensifs en recherche et développement, qui requièrent dès le départ des financements massifs et risqués. La bonne échelle, c'est donc l'échelle européenne. Pour répondre à cet impératif, le Président de la République a proposé la création d'une agence européenne pour l'innovation de rupture. Nous ne pouvons pas prendre de retard. Dès 2019, un prototype d'agence doit être mis en place au niveau européen. Enfin, nous devons saisir le tournant de l'intelligence artificielle. Au niveau national, d'abord, où c'est une priorité avec le déploiement de 1,5 milliard d'euros en cinq ans, mais surtout avec un programme très structuré. En Europe, ensuite, en soutenant la stratégie formulée par la Commission européenne, en particulier sur les trois axes proposés : la compétitivité technologique et économique ; l'anticipation des changements socio-économiques ; la création d'un cadre juridique et éthique.

Deuxième point : nous voulons une Europe ouverte, mais également capable de défendre ses valeurs, ses intérêts et son modèle économique. Il est absolument nécessaire de défendre des relations commerciales ouvertes et réciproques, à l'heure où se développent des pratiques commerciales déloyales et la tentation du protectionnisme. Nous devons agir fermement, dans le respect du droit, pour défendre, moderniser et renforcer les règles du commerce international et permettre ainsi à nos entreprises d'évoluer dans un environnement sûr et favorable à l'innovation et aux investissements. Mais ouverture ne signifie pas naïveté ; nous voulons aussi nous protéger lorsque des pays tiers ciblent, de façon parfois agressive, des entreprises stratégiques en Europe. C'est pourquoi nous devons adopter rapidement le règlement sur le filtrage des investissements étrangers en Europe. S'agissant des enjeux nouveaux liés à l'économie numérique, l'Europe doit proposer un modèle juste et efficace. Elle a su le faire en matière de protection des données personnelles. Il faut avancer sur deux autres défis qui sont posés. D'une part, sur la fiscalité : il n'est pas acceptable que les grandes entreprises du numérique ne paient que 9 % d'impôts en Europe, contre 23 % pour les acteurs traditionnels. C'est vrai ! C'est non seulement injuste, mais aussi dangereux pour notre compétitivité et pour nos finances publiques. D'autre part, sur la concurrence : c'est un fait, les distorsions de concurrence existent pour les plateformes qui n'ont pas les mêmes obligations réglementaires, sociales et fiscales. Nous sommes déterminés à contrôler et à sanctionner les pratiques déloyales, car il faut assurer la juste concurrence et des relations commerciales équilibrées entre les acteurs économiques. Nous le faisons sur le plan national. En mars dernier, Bruno Le Maire a assigné Google et Apple en justice pour pratiques commerciales abusives, comme il l'avait fait contre Amazon en 2017. Nous portons ces principes au sein de l'Union, où nous voulons une régulation européenne des relations d'affaires des plateformes avec leurs partenaires. La France s'est mobilisée pour que la Commission européenne propose un tel encadrement, nous soutenons entièrement le projet déposé le 26 avril dernier, en particulier la mise en place d'un observatoire européen sur la loyauté des plateformes numériques. Ce projet doit aboutir.

nous voulons une Europe qui défend ses intérêts, une Europe qui met au coeur de ses projets la compétitivité et l'industrie, une Europe qui se positionne avec force sur les grands enjeux technologiques d'avenir. Voilà les grands messages que je souhaitais vous adresser en ouverture de ce débat. Je me ferai un plaisir de préciser tous ces points en répondant à vos questions.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des affaires européennes, mes chers collègues, au sommet de Tallinn du 29 septembre 2017, il a été décidé de faire de l'Europe un chef de file au niveau mondial dans le domaine du numérique. Le Conseil européen du 19 octobre a acté cette volonté partagée par tous les États membres. Dans ses conclusions, le Conseil a énuméré un certain nombre de chantiers à ouvrir ou à approfondir dans la perspective de l'Europe numérique. Parmi ceux-ci, je veux évoquer en particulier celui de l'approche commune de la cybersécurité. Comme l'a rappelé Jean-Claude Juncker dans son discours sur l'état de l'Union, « les cyberattaques sont parfois plus dangereuses pour la stabilité des démocraties et des économies que les fusils et les chars ». En effet, la lutte contre les cyberattaques représente un défi majeur. En 2016, on a recensé 4 000 attaques par rançongiciel chaque jour et 80 % des entreprises européennes ont été touchées par au moins un accident lié à la cybersécurité. Au regard de la rapidité des évolutions technologiques et de l'ampleur du défi, il y a urgence à agir et à mobiliser les moyens. Aux États-Unis, l'investissement consacré à la cybersécurité est quatre fois plus élevé qu'en Europe. La commissaire européenne à l'économie et à la société numériques a demandé un doublement

Par ailleurs, l'Union européenne envisage de transformer l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information en véritable agence de cybersécurité de l'Union. Le rôle de cette nouvelle agence serait d'aider les États membres, les institutions de l'Union européenne et les entreprises à contrer les cyberattaques. Sachant que la France dispose déjà de la solide Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, comment va s'articuler le rôle de l'agence européenne avec notre agence nationale ? La parole est à Mme la secrétaire

de révision du mandat de l'ENISA, l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, comme vous l'avez mentionné, la création d'un centre de compétences et de recherche européen sur la cybersécurité, ainsi qu'une proposition pour une réponse coordonnée lors d'incidents et de crises de cybersécurité de grande échelle.

Nous nous félicitons, par ailleurs, du choix de l'Union européenne de mettre en place en son sein un outil utilisé par plusieurs États membres précurseurs depuis près de vingt ans- la certification de sécurité -, qui sera un élément-clé pour renforcer la sécurité et la confiance dans le numérique au sein de l'Union. Dans les négociations sur la certification, la France veillera à ce que l'échelon européen garantisse une harmonisation des niveaux de sécurité, en préservant, pour les hauts niveaux de sécurité, d'une part, la réalisation d'expertises réalisées par des tiers indépendants et, d'autre part, le rôle des États. Enfin, la France soutient l'idée de renforcer les missions de l'ENISA. Cette dernière doit avoir une véritable valeur ajoutée au niveau européen en tant que soutien aux États membres dans l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques liées à la cybersécurité ou par le partage et l'accès à des informations et analyses à l'état de l'art, tout en respectant les compétences techniques et opérationnelles des États membres. La parole

continent. En France, même si l'investissement des entreprises et des collectivités territoriales en matière de recherche et développement a progressé au cours des dernières années, on constate cependant un recul de la situation relative de notre pays à l'échelle internationale tant la compétition à laquelle se livrent les pays asiatiques, mais aussi les autres pays européens et des pays développés, est forte en la matière. En 2016, on ne comptait qu'une trentaine d'entreprises françaises parmi les 1 000 entreprises mondiales investissant le plus en recherche et développement. L'enjeu est donc considérable en termes tant de compétitivité de notre industrie que de création d'emplois. Cela fait partie de la vision nationale

Où en sommes-nous dans la mise en place de notre stratégie dans ce domaine au moment où la Commission européenne vient de présenter ses premières propositions pour le cadre pluriannuel financier 2021-2027 ? Où en est-on également dans la concrétisation, vous l'avez évoqué,

Par ailleurs, dans l'attente de la création de cette agence à l'échelle européenne, la France entend-elle créer une agence nationale de ce type en renforçant, par exemple, les missions et les moyens alloués à l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ? La parole

pour commencer à agir : nous travaillons avec la Commission sur la préfiguration de cette initiative et sur la possibilité de mettre en route des actions dès 2019. Nous avons formulé des suggestions concrètes afin que les caractéristiques-clés de la proposition du Président de la République- des financements élevés, une forte prise de risque, un management agile -figurent dans le projet pilote. un instrument qui soit, à terme, entièrement européen et pas limité à quelques États membres, car une telle initiative est appelée à contribuer au technologique de l'ensemble de l'industrie européenne. En outre, cette initiative requiert une masse critique de financements qui ne peut être atteinte qu'à l'échelon européen.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, chers collègues, le développement des technologies, qui transforment en données numériques nos comportements et nos relations avec les entreprises et les administrations, nous impose de veiller avec la plus grande vigilance à la défense des libertés individuelles. auquel vous appartenez, madame la secrétaire d'État, a pris des engagements dans ce domaine, notamment en garantissant aux citoyens l'impossibilité d'une automatisation complète des décisions individuelles prises par l'administration. Je rappelle que la directive européenne relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel nous y oblige. Lors de la discussion au Sénat du projet de loi ayant pour objet sa transposition, la Haute Assemblée, à l'unanimité, a été troublée par les libertés prises par votre gouvernement avec les principes forts de la directive, notamment en ce qui concerne la dérogation accordée aux établissements universitaires de mettre en oeuvre des traitements automatisés des informations personnelles collectées par la plateforme Parcoursup. Un grand quotidien du soir vient d'apporter les preuves de ce que le Sénat soupçonnait : ces traitements sont massifs et certaines universités utilisent même des logiciels de classement automatique des dossiers qui leur sont fournis par votre gouvernement. Le 12 avril dernier, le Sénat, à l'unanimité, je le répète, sur proposition de sa commission des lois et de sa rapporteur, Mme Sophie Joissains, a défendu une rédaction de ce texte qui protège les droits individuels, conformément à l'esprit de la directive européenne.

que l'Europe pourra construire son approche, son modèle, afin de protéger ses valeurs, pour peser et d'être plus influente dans le développement de l'utilisation de ces technologies. Ce cadre, qui est un élément clé, me semble au contraire extrêmement positif et extrêmement favorable au développement des technologies de type intelligence artificielle

de prendre prouvent que vous êtes d'accord avec la position du Sénat, ce dont je me félicite. Vous allez donc mettre en oeuvre pour la dernière lecture de cette loi à l'Assemblée nationale une transposition de l'esprit même de la directive, comme le réclame

en mars dernier, cinquante entreprises de dix-neuf États membres de l'Union européenne ont appelé les décideurs politiques européens et nationaux à revoir le projet de règlement « e-Privacy Elles s'alarment des dispositions envisagées au niveau européen qui, selon elles, n'offriront pas une protection efficace des citoyens, nuiront au développement de l'économie numérique européenne et porteront atteinte au rôle essentiel des médias dans la vie démocratique, tout en renforçant les positions des acteurs déjà dominants de l'économie de la donnée et en privant les acteurs numériques européens de relations directes et de confiance avec les utilisateurs de leurs services. En France, suite au rapport Villani, nombre d'entreprises s'interrogent sur la manière dont l'usage de l'intelligence artificielle va être encadré. Ces dispositions, vous le savez, madame la secrétaire d'État, détermineront leur champ de travail et leur compétitivité à l'égard de concurrents étrangers, comme la Chine et les qui exploitent les données de leurs citoyens sans réelles contraintes. Le rapport de Cédric Villani met également en avant les capacités importantes de la France en matière de recherche sur l'intelligence artificielle. De fait, de grandes entreprises américaines et asiatiques implantent des laboratoires de recherche sur le Il est donc essentiel, madame la secrétaire d'État, que vous précisiez la position éthique qui sera celle de la France au sujet de l'intelligence artificielle, tant en amont, dans la collecte et le traitement des données des citoyens, qu'en aval, sur les relations entre intelligence artificielle et être humain.

les sujets éthiques, qui sont extrêmement prégnants dans nos discussions, au niveau français comme au niveau européen.

d'ici à 2020 et de le porter ainsi à 20 milliards d'euros, la Commission souligne que l'Union européenne et les États membres devront orienter leurs ressources vers des secteurs stratégiques : la santé, l'environnement et les mobilités. De plus, afin d'éviter toute dilution des moyens, qui s'apparenterait à une gabegie, la Commission prône une coordination à l'échelle européenne des politiques menées par les États membres. Dans cette perspective, quelle est la position du Gouvernement sur l'idée d'un fonds commun européen

Notre assemblée a ainsi adopté une résolution sur le règlement concernant un cadre applicable à la libre circulation des données à caractère non personnel dans l'Union européenne, exprimant des doutes sur sa pertinence et s'étonnant que ledit règlement ne définisse même pas

secrétaire d'État. Madame la sénatrice, l'intelligence artificielle ne sera compétitive en Europe que si elle a accès au plus grand nombre de données.

devenue un point focal de préoccupation des consommateurs. La CNIL a d'ailleurs souligné que la collecte disproportionnée de données personnelles faisait partie des craintes les plus partagées concernant les algorithmes. algorithmes. Nous souhaitons avoir l'opportunité de faire émerger un écosystème vertueux qui puisse devenir un réel facteur de différenciation et de compétitivité pour les entreprises européennes dans le cadre du RGPD. Un autre atout de l'Europe, c'est la richesse de ses gisements de données. On résume souvent les batailles industrielles dans le domaine de l'intelligence artificielle à la seule question des données, en faisant allusion à l'avance prise par les géants de l'internet.

L'intelligence artificielle peut être alimentée par une grande diversité de données, qu'elles soient industrielles, environnementales, médicales, juridiques ou liées aux services publics, données sur lesquelles l'avantage est parfois favorable aux acteurs européens. Enfin, le marché unique numérique, qui offre un cadre protecteur et harmonisé au niveau européen, constitue un facteur de compétitivité de long terme. S'agissant des moyens que vous avez mentionnés, nous nous félicitons que la Commission européenne soutienne la recherche et le développement en matière d'intelligence artificielle. En effet, dans sa proposition du 25 avril dernier figure l'annonce d'une augmentation de l'investissement public dans le cadre d'Horizon 2020 de 1,5 milliard d'euros pour la

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, grand défi de ce XXI siècle, l'intelligence artificielle est aujourd'hui déjà un enjeu diplomatique de premier plan. Dans la course entre la Chine et les États-Unis, la France seule ne peut rivaliser avec ces géants étrangers. Elle a besoin d'être épaulée par l'Europe. Preuve en sont les 20 milliards dépensés par la Chine en 2016 pour financer le développement de l'intelligence artificielle, quand notre pays peine à dégager une enveloppe de 1,5 milliard d'euros. L'effort du Président de la République mérite d'être salué, mais il n'est pas suffisant. À la fin du mois de mars 2018, le mathématicien et député Cédric Villani a dressé une liste de recommandations pour assurer le développement de l'intelligence artificielle aux niveaux national et européen mise à disposition des données publiques sur l'agriculture, l'énergie, la météo ou le climat dès 2019, facilitation des expérimentations numériques, avancées sur la transformation du travail ou encore création d'un réseau d'instituts interdisciplinaires de recherche sur l'intelligence artificielle. L'appel français a été entendu. Le 10 avril dernier, vingt-quatre États membres, plus la Norvège, ont signé une déclaration commune de coopération sur le sujet, assurant que ces défis numériques devaient être relevés collectivement.

du projet de supercalculateur européen dédié aux applications de l'intelligence artificielle, que le rapport Villani appelait de ses voeux ? secrétaire d'État. Madame la sénatrice, vous mentionnez les efforts à faire en matière de recherche et développement. Il s'agit bien, en effet, du premier axe de la stratégie française en matière d'intelligence artificielle annoncée par le Président de la République : il faut former et attirer les meilleurs chercheurs pour rester à la pointe de la compétition mondiale et permettre l'émergence de futurs champions industriels.

des meilleurs chercheurs internationaux par le lancement d'un programme de chaires individuelles internationales et nationales. Enfin, des appels à projets de recherche en innovation de rupture seront lancés. Voilà ce qui sera fait au niveau français, en plus de l'assouplissement proposé de la loi Allègre, afin de permettre des allers-retours et une fructification croisée entre le monde de l'entreprise et celui de la recherche. La Commission européenne, quant à elle, accompagne également également fortement la recherche et le développement en matière d'intelligence artificielle, avec le soutien à l'émergence et au renforcement des centres de recherche d'excellence en intelligence artificielle, l'encouragement à la collaboration européenne et le soutien aux expérimentations, notamment celles qui s'appuient sur les pôles d'innovation numérique. La parole

L'intelligence artificielle pourra certainement aider à la décision sur de nombreux sujets, comme le choix des implantations, la fourniture d'une meilleure irrigation, tout en en apportant des améliorations en matière environnementale. Outre-Atlantique, les agriculteurs disposent d'ailleurs déjà d'un certain nombre d'outils d'intelligence augmentée. L'Europe dispose d'importants atouts à faire valoir dans ce domaine, mais je crains qu'elle ne soit déjà quelque peu dépassée par les GAFA. Ma question porte donc sur les moyens mis en oeuvre par l'Union européenne pour saisir ces nouvelles perspectives en matière d'agriculture. Dans ce domaine, nous avons le droit de temps en temps de parler un peu de modernité et pas que de passéisme La Commission européenne envisage-t-elle, par exemple, une application de l'intelligence artificielle à la définition des zones à contraintes spécifiques ? Je veux parler plus particulièrement des zones défavorisées.

qu'il est aujourd'hui appelé à faire face à des défis de plus en plus importants, afin de garantir au plus grand nombre une alimentation saine, abordable et respectueuse de l'environnement. Les états généraux de l'alimentation ont montré la sensibilité des consommateurs et des citoyens à ces questions. L'intelligence artificielle peut apporter des solutions au double défi de la compétitivité et du respect de l'environnement. Les outils numériques permettant d'assister l'agriculture dite « de précision » sont déjà largement utilisés et de nombreuses start-up françaises réinventent les services aux agriculteurs Naïo Technologies et ses robots agricoles autonomes, Airinov et ses capteurs connectés, Carbon Bee AgTech et ses caméras intelligentes pour détecter les maladies, et j'en passe Cet écosystème est donc foisonnant, et l'enjeu est désormais de le transformer en une véritable filière. Les défis de court terme que nous voyons sont aujourd'hui de deux types. de la construction des infrastructures essentielles, avec la couverture réseau des exploitations, le soutien à la recherche et à l'innovation en matière de robotique et d'objets connectés et les enjeux liés aux données- leur interopérabilité, leur propriété et la loyauté de leur utilisation. Le deuxième enjeu est de former les agriculteurs et de les préparer, ainsi que l'ensemble de leur écosystème, à ce nouveau paradigme. Les métiers se transforment profondément, avec une demande renforcée en matière de transparence, de traçabilité et de circuits courts. Cela ouvre des perspectives importantes. Je note également votre suggestion relative à l'utilisation de l'intelligence artificielle en matière de zonage,

Ce même rapport pointe le risque pour la France de se faire distancer rapidement par les entreprises américaines et asiatiques. C'est malheureusement déjà le cas ! Si le président Emmanuel Macron a déclaré vouloir faire de la France une « », force est de reconnaître qu'aujourd'hui les moyens ne suivent pas. Devant les investissements massifs de nos concurrents, le modeste fonds pour le financement de l'innovation, lancé à grands renforts médiatiques par le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, ne pèsera pas bien lourd avec ses 200 millions d'euros de dotation annuelle. Même réalité navrante, lorsque l'on constate que l'État, incapable de respecter financièrement les délais initiaux, décale à 2027 la livraison de la ligne 18 du Grand Paris Express, pourtant indispensable à la déserte du plateau de Saclay. Je rappelle au passage que l'ambition de départ était de créer « la » Silicon Valley européenne ... Je crains qu'elle ne le devienne à la fumée des cierges ! Dans ces conditions, mes chers collègues, comment la France peut-elle devenir une, un exemple pour l'Union européenne ? sur l'innovation la France propose-t-elle à l'Europe pour attirer les jeunes générations ? Les entrepreneurs de la French Tech ont démontré leur savoir-faire et leur dynamisme. L'État doit maintenant faire sa part en accompagnant efficacement ceux qui sont prêts à prendre des risques. L'Europe aussi doit voir ces nouvelles technologies comme une chance pour l'avenir. Par exemple, à quand un MIT européen, emblématique d'une politique commune ? L'Europe doit être conquérante ! Le risque est de voir l'avenir s'écrire sans elle, et donc sans nous. La France peut, et doit, être une locomotive européenne. Quels moyens, madame la secrétaire d'État, entendez-vous réellement y consacrer ? secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, je vous remercie de votre question. On constate en effet qu'un duopole Chine-États-Unis est en train d'émerger au niveau mondial. Au niveau européen, la France est au coude à coude avec le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Suisse en matière de force de frappe de recherche et d'expertise. S'agissant des publications de recherche, notre pays se situe dans le peloton de tête au niveau mondial, au coude à coude avec le Canada, mais toujours derrière le duopole Chine-États-Unis. En ce qui concerne l'innovation, la France occupe un rang moyen. L'investissement dans les start-up d'intelligence artificielle est deux fois moindre qu'au Royaume-Uni. La Chine, dans ce domaine, est en train de dépasser les États-Unis. Ainsi, 48 % des 15 milliards de dollars investis dans les start-up de l'intelligence artificielle dans le monde en 2017 sont allés à la Chine et 38 % aux entreprises américaines.

Il faut donc compter sur nos atouts, que j'ai déjà eu l'occasion d'énumérer. Je les rappelle, il s'agit du cadre précurseur et exigeant que nous avons en matière de protection des données personnelles, qui constitue un véritable avantage compétitif pour nos entreprises si elles s'en emparent, du gisement des données, en particulier des données structurées qui peuvent avoir une grande valeur pour l'intelligence artificielle, et du marché unique numérique. Par ailleurs, nous investissons fortement dans l'innovation de rupture, et une partie de cet investissement ira à l'intelligence artificielle. Nous avons annoncé

à créer l'entreprise commune qui portera l'ambition européenne en la matière, avec la volonté d'investir dans des machines exaflopiques,

l'Union européenne que le Président de la République et le Gouvernement souhaitent construire est un espace intégré qui permet de développer des politiques qui sont mieux traitées à cet échelon qu'à celui des États. Cette volonté de redéfinir finalement la subsidiarité, nous la partageons. Il convient de définir les matières retenues et d'afficher des ambitions fortes.

En matière de politique numérique et de télécommunications, chaque État a développé aujourd'hui ses propres règles juridiques. Certains règlements européens sont les bienvenus ; néanmoins, une plus grande intégration peut et doit avoir lieu. Ainsi, pourriez-vous nous dire si les négociations sur une forme de code européen des communications électroniques avancent ? Si oui, à quelle échéance ? Comme en matière fiscale, il ne faudrait pas de dumping entre nous, qui créerait une concurrence qui affaiblirait chacun. Une autre question importante concerne les outils de régulation. Ensuite, en matière d'aménagement, qu'en est-il du déploiement de la 5G dans notre pays ? Le monde s'y prépare, comme une nouvelle révolution numérique. Cependant, les degrés actuels d'engagement des pays varient énormément, qui aura des conséquences fondamentales sur le développement économique, en particulier avec l'essor de la notion d'internet des objets. Les États vont devoir choisir entre les rentrées d'argent liées à l'attribution de fréquences à des tarifs élevés

sur la couverture 5G en Europe. Il s'agit en effet d'éléments de capacité qui sont extrêmement importants pour que notre continent soit en pointe en matière d'innovation et de numérique. S'agissant de la régulation de l'accès aux réseaux de communications électroniques, la négociation est aujourd'hui bloquée entre le Conseil et le Parlement. Le trilogue du 25 avril dernier a été un échec sur ce point. Les termes du débat n'ont pas sensiblement évolué par rapport à la présentation faite dans la note. Nous tentons de préserver l'équilibre actuel du cadre réglementaire de la fibre et les marges de manoeuvre du régulateur. En ce qui concerne la réglementation des services de communications électroniques, la négociation a permis de conserver le principe de l'extension du champ du paquet télécom aux services OTT,, c'est-à-dire les services de type WhatsApp, qui se superposent Quant à la 5G, c'est une nouvelle technologie pour les réseaux mobiles au service de la numérisation de notre industrie et de notre économie. Elle apportera plus de capacité avec moins de latence et davantage de sécurité en consommant moins d'énergie. C'est donc un enjeu stratégique pour l'industrie, la compétitivité, l'innovation et les services publics rénovés. Elle facilitera, voire permettra, le développement des transports autonomes, de la télémédecine, de la ville intelligente, de l'usine du futur et de la réalité augmentée. Au niveau européen, la Commission a détaillé, dans une communication de septembre 2016, un premier plan d'action et demande à chaque État membre d'en élaborer un au niveau national. Les États membres sont encouragés à établir une feuille de route en vue d'une introduction de la 5G d'ici à la fin de 2018 et d'un déploiement commercial en 2020. Sur ce point, nous travaillons avec l'ARCEP, pour lancer les expérimentations qui permettront à la fois de tester les technologies, mais aussi de voir grandeur nature comment développer des modèles d'affaires autour de cette nouvelle technologie sur notre territoire. La parole

Je veux y croire, car je suis également préoccupé par la défense de nos données personnelles. Toutefois, nous devons aussi être méfiants. aussi être méfiants. Je reviens de Chine, et je constate qu'il est probable qu'un certain nombre d'innovations technologiques majeures, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle, se feront sur la base de données qui n'auront pas nécessairement été collectées dans le respect de nos principes éthiques. Il est aussi probable que ce type de pratiques conduise à apporter à certains pays n'ayant ni

à terme, la manière dont nous pourrons maîtriser l'évolution des technologies, nos données et les capacités de nos entreprises à être

souhaitons faciliter l'accès aux données pour des motifs de recherche et d'innovation dans trois directions : du public vers le privé, du privé vers le public et entre acteurs privés. D'abord, il s'agit d'ouvrir un débat sur l'accès aux bases de données des monopoles de fait que constituent les grandes plateformes. il s'agit de lancer des appels à manifestation d'intérêts pour la création de plateformes de partage de données entre acteurs, par secteur ou intersecteurs, ce qui permettrait d'associer des données en provenance du secteur public et du secteur privé.

Madame la secrétaire d'État, depuis septembre 2015, l'Union européenne investit pour relancer l'industrie. Initialement prévu jusqu'en 2018, ce plan d'investissement, ou plan Juncker, a été conforté jusqu'à l'horizon 2020 avec un objectif de financement porté à 500 milliards d'euros grâce à l'effet de levier. Par l'intermédiaire du Fonds européen pour les investissements stratégiques, les projets les plus prometteurs, mais aussi les plus risqués, trouvent une source de financement. Pour être financé par ce fonds, un projet doit s'inscrire dans un des sept secteurs prioritaires, parmi lesquels le développement et le déploiement des technologies de l'information et de la communication » ou encore « la promotion du capital humain, de la culture et de la santé ». Depuis plusieurs années déjà, avec l'organisation de la semaine européenne des compétences numériques en mars 2012, la Commission européenne a conscience que les technologies numériques sont stratégiques, voire vitales, pour les économies du XXI siècle. Depuis 2013 existe une semaine européenne du code, dont la prochaine édition aura lieu du 6 au 21 octobre 2018. Lors de la dernière édition en 2016, près de 970 000 participants issus de cinquante pays ont pris part à plus de 23 000 événements. En décembre 2016, la Commission lançait la coalition en faveur des compétences et des emplois dans le secteur du numérique pour aider les Européens dans leur parcours professionnel et leur quotidien. À cette occasion, Günther Oettinger, à l'époque commissaire européen à l'économie et à la société numériques, a fait valoir que « le manque de compétences numériques constitue déjà un frein à l'innovation et à la croissance en Europe. Pas seulement pour les entreprises du secteur des TIC, mais aussi pour les organisations dans tous les secteurs- tant privé que public. » Dans le domaine du numérique, les investissements concernent aujourd'hui essentiellement le déploiement du très haut débit, à l'exemple du projet porté par la région Grand Est.

plus recherchés. Comment aujourd'hui mieux orienter les crédits du Fonds européen pour les investissements stratégiques vers des actions immatérielles, notamment le développement des compétences numériques comme le codage, qui préparent la compétitivité future des économies européennes ? Comment redonner la main aux États membres alors que, dès 2014, des grandes entreprises comme Microsoft ou Facebook ont lancé une initiative européenne pour le codage ?

pour accélérer la formation numérique des jeunes ou des personnes éloignées de l'emploi, afin de mettre les choses en place extrêmement rapidement. Je suis d'accord avec vous, la formation et la constitution de compétences

En effet, dans son discours sur l'état de l'Union en septembre 2017, il affirmait que « les cyberattaques sont parfois plus dangereuses pour la stabilité des démocraties et des économies que les fusils et les chars ». 2017 a été marquée par la succession de cyberattaques de plus en plus professionnelles et sophistiquées, qui ont ébranlé la sécurité des citoyens, des entreprises et parfois même des États.

Le numérique est incontestablement un vecteur d'innovation et de croissance, mais il crée des poches de vulnérabilité. La cybermenace s'intensifie au rythme de la numérisation du monde, et toute entreprise est une cible potentielle.

Il est ainsi urgent de constituer un front commun pour protéger le savoir-faire industriel européen des cyberattaques internationales et investir massivement dans la sécurité, sous peine d'une perte totale de confiance dans l'outil numérique. Afin d'intensifier la coopération entre les États membres, une première directive européenne a été adoptée en 2016, la directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, ou SRI, transposée dans le droit français le 15 février 2018. La Commission européenne a par ailleurs proposé en septembre 2017 un paquet cybersécurité, qui vise à instaurer un système européen de certification du niveau de cybersécurité des produits technologiques, à réformer l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information,

la cybersécurité est-elle, selon vous, une question de souveraineté nationale ou européenne et comment faire de la sécurité en matière numérique un facteur de compétitivité pour l'Europe et un avantage concurrentiel pour les entreprises françaises ? La parole est à Mme la

: cette directive, dont la date limite de transposition était aujourd'hui, et le paquet cybersécurité de septembre 2017, qui apportera des éléments importants importants sur la révision du mandat de l'ENISA, sur la création d'un centre européen de compétences et de recherche et sur l'élaboration d'une réponse coordonnée aux incidents et aux crises de cybersécurité

avec une vigilance sur la souveraineté nationale. En effet, il y a, dans les technologies de cybersécurité et dans les données que celles-ci protègent, des éléments de souveraineté nationale.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, tous les observateurs sont d'accord sur au moins un point : depuis quelques années, l'intelligence artificielle est entrée dans une nouvelle ère. Elle est devenue l'une des technologies les plus stratégiques, susceptible d'initier une véritable révolution industrielle et technologique- nous avons tous en tête ces mots de Vladimir Poutine, selon lequel « celui qui deviendra dans ce domaine maîtrisera le monde il s'y connaît ... Aux côtés des États-Unis et de la Chine, incontestablement très en avance, le Canada, le Royaume-Uni et Israël sont également fortement mobilisés pour développer de nouvelles applications, notamment dans les secteurs de la santé et de l'automobile. Il est grand temps que l'Europe prenne toute sa place dans ce défi majeur et, compte tenu du Brexit, la France doit jouer, aux côtés de l'Allemagne, un rôle moteur dans l'élaboration d'une stratégie européenne. Dans ce contexte, je me réjouis de l'ambition affichée par le président Emmanuel Macron le 29 mars dernier corroborée par le gouvernement allemand, qui prévoit notamment la création d'un centre commun d'intelligence artificielle avec la France. Toutefois, pour ne pas rater ce virage, les investissements

De même, la mise en place de chaires individuelles et la modification de la réglementation concernant la recherche vont incontestablement dans le bon sens. Cela dit, la préconisation du rapport Villani visant à revaloriser de manière très significative le salaire des chercheurs, notamment en tout début de carrière, est un paramètre essentiel dont le Président de la République n'a visiblement pas voulu tenir compte. C'est très regrettable, et je ne peux me satisfaire de constater que nos talents quittent massivement et irrémédiablement la France et, plus largement, l'Europe, pour rejoindre la Silicon Valley.

secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, ce que nous souhaitons avant tout, c'est faire valoir les atouts de la France et de l'Europe en matière d'intelligence artificielle et l'excellence de la recherche française dans les domaines scientifiques et technologiques- les mathématiques, l'informatique, les sciences des données

Le Gouvernement a mis en place de nombreuses actions de soutien en faveur de la R&D, d'une part, et de l'émergence et du développement des start-up, d'autre part. Au sein du fonds pour l'innovation de rupture, il y aura un compartiment dédié financement de projets dits de « », dont une partie sera consacrée à l'intelligence artificielle. Il s'agit vraiment d'initiatives qui doivent être pilotées et recentrées, et non d'un saupoudrage ou d'un redéploiement de façade. Il y a donc une véritable volonté d'aligner les moyens avec les enjeux. Je rappelle aussi que la France compte de grandes entreprises de services dans le numérique, qui vont être clés pour mener à bien cette stratégie- Capgemini, Atos ou encore Sopra Steria -, et ces entreprises investissent dans les technologies d'intelligence artificielle. Enfin, de très grands groupes français utilisateurs de technologies sont aussi des références dans leur secteur

d'éléments exploitables pour faire en sorte que l'on joue pleinement notre partition dans ces enjeux de l'innovation et de l'intelligence artificielle. La parole

cette chambre à une culture d'avenir, et la digitalisation de l'économie et l'intelligence artificielle ne lui sont pas étrangères. Je rappelle que, le 21 juin prochain, nous assisterons à la restitution d'un rapport spécifique

cette évolution de l'économie et de la compétitivité de l'Union européenne marquera le développement du marché unique, un des grands joyaux de la création de l'Union européenne.

Le marché unique européen est quelque chose que nous devons protéger avec la plus grande vigilance, parce que c'est notre atout dans la compétition internationale. C'est également notre atout dans le cadre des négociations commerciales internationales.

le concept d'extraterritorialité des lois américaines. Depuis 1996, l'Union européenne est dotée des mêmes outils pour faire valoir l'extraterritorialité des lois européennes ; simplement, il n'y a pas de volonté politique de notre principal partenaire, l'Allemagne, en la matière. Nous devons mettre en place cette extraterritorialité des lois européennes, non pas pour assouvir une quelconque vengeance, mais tout simplement parce que l'Union européenne doit, au travers de cela, marquer sa puissance. Enfin, nous souhaiterions mettre en

Si quelques pays, notamment la France et l'Allemagne, peuvent avancer et montrer le chemin à d'autres États, nous aurons été dans l'esprit européen. Je signale en outre que ce sera seulement à la fin de cette